La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre III.

ou encore en mission temporaire, en apprentissage ou en stage, est, comme l'ont fait remarquer la Fondation Abbé Pierre et le Défenseur des droits, un bail de précarisation des précaires. En tant que bail non renouvelable d'une durée maximale de dix mois et non soumis aux protections de la loi du 6 juillet 1989, il forme le terreau favorable à des situations dans lesquelles les locataires seraient contraints d'aller de bail court en bail court.

pour les précaires. Si créer une offre locative adaptée à ce type de publics peut être un objectif louable- cela répond à une demande de la part des locataires et des propriétaires en revanche, c'est l'absence de mesures visant à éviter une pérennisation de ces baux mobilité au détriment des baux meublés classiques qui, pourtant, garantissent une plus grande sécurité aux locataires. En effet, les propriétaires trouveront un avantage évident à louer leurs biens en bail mobilité, puisque ce type de bail bénéficie du dispositif VISALE, ou visa pour le logement et l'emploi, qui garantit le paiement des loyers et des charges et la remise en état du logement en cas de dégradation. De surcroît, le loyer peut être fixé librement par le propriétaire. Augmenter la mobilité des locataires sans leur garantir un logement au terme du contrat de location, c'est comme flexibiliser le marché du travail sans renforcer la sécurité : c'est précariser les plus fragiles et les plus vulnérables. En outre, l'utilisation de la notion de « mission temporaire » dans l'énumération des publics visés par le bail mobilité peut mener à la confusion. Qu'est-ce qui est temporaire ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé destiné aux personnes qui suivent une formation professionnelle, des études supérieures, sont en contrat d'apprentissage, en stage, en service civique ou en mission professionnelle.

véritable fléau des centres-villes des grandes villes. Le bail mobilité permettra en effet de louer le logement en basse saison à des étudiants ou à des actifs en mobilité,

On le sait, la location temporaire est bien plus lucrative que la location classique, et bien moins contraignante. Ces outils de location vont aggraver la tension sur le marché, détourner des logements supplémentaires du parc locatif classique et contribuer à l'augmentation des loyers, notamment dans les grandes villes et dans les villes très touristiques. Par ailleurs, toutes les mesures protectrices d'ordre public du locataire s'appliquent uniquement si le logement est la résidence principale du locataire. Celui qui ne dispose pas d'un autre logement sera inévitablement mis en difficulté à la fin du bail ; la mobilité devient alors forcée.

Je voterai ces amendements de suppression. Je suis convaincue que le bail mobilité n'est pas la bonne solution au problème du logement des jeunes en stage.

? La tradition du droit sur les baux en France est justement de scinder ce qui relève d'une résidence principale de ce qui relève des activités commerciales.

est une des conditions d'émancipation, d'autonomie et d'indépendance de celui qui sort de

formules diverses de logements puissent être mises en place, à côté notamment du logement familial. Je pense à la possibilité de se loger dans des conditions plus souples sur un lieu ou sur différents lieux d'activité professionnelle. Le public qui a été ciblé comme pouvant

et l'amélioration de la péréquation entre les bailleurs de ce parc. Enfin, il est prévu de réformer le cadre fiscal de l'investissement locatif privé, avec notamment le remplacement du dispositif Pinel par un régime de déduction des charges de propriété pour l'ensemble des investisseurs.

Or changer d'emploi est souvent synonyme de changement de ville. Les personnes en mutation professionnelle manquent de point d'appui et ne peuvent pas forcément s'engager dans un bail traditionnel. La flexibilité offerte par le bail mobilité permet de répondre à cette difficulté et d'accompagner ces changements de vie, parfois très difficiles. L'amendement s'inscrit ainsi pleinement dans la philosophie du texte qui vise, notamment, à lutter contre « l'assignation à résidence » en offrant à chacun la possibilité de vivre et d'évoluer en fonction de ses besoins.

dans l'attente du déménagement de l'ensemble du ménage et d'une installation plus durable. Ouvrir le champ du bail mobilité aux salariés en mutation professionnelle est de nature à offrir une solution de logement supplémentaire à ces personnes pour lesquelles la mobilité constitue un point d'appui dans le parcours professionnel.

J'ai expliqué tout à l'heure qu'une de mes craintes était qu'on entre dans un mécanisme qui finira par modifier les fondamentaux du droit s'agissant des garanties données aux résidences principales.

mon collègue Xavier Iacovelli pourrait en faire autant -de l'expérience d'un sénateur dans un département où la pression foncière est absolue. Dans un département comme le nôtre, les droits ne sont jamais du côté du locataire, ils

si vous êtes des propriétaires citoyens, remettez votre logement sur le marché de la location, y compris en passant par une association agréée d'intermédiation locative. Il n'en reste pas moins que certains propriétaires

Le caractère dérogatoire du bail mobilité est un recul en termes de garanties et de droits pour les locataires, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler. Le Défenseur des droits a d'ailleurs souligné que « la protection réduite des droits du locataire et la libre fixation du loyer qui sera inéluctablement tiré à la hausse dans un contexte de concurrence avec les locations touristiques de courte durée comme le montre l'étude d'impact, expose finalement le public visé, principalement des jeunes, à une précarisation accrue de leurs conditions d'accès au logement C'est pourquoi notre amendement de repli vise à éviter que le bail mobilité ne devienne un passe-droit des marchands de sommeil, qui y verraient l'occasion de continuer à encaisser des loyers au prix fort, pour un logement non décent, voire insalubre ou dangereux, en évitant la procédure de suspension ou de réduction du loyer, instituée par l'article 20-1 de la loi de 1989, et applicable aussi bien aux locations nues du titre I, qu'aux locations meublées visées par le titre I de la loi de 1989.

par les commissions départementales de conciliation, particulièrement efficace, évite le recours à un juge. Certes, le bail mobilité induira moins de contentieux que les baux classiques en l'absence de dépôt de garantie ou de la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire. Cependant, le recours à ces commissions n'est pas superflu dans le cadre d'un bail mobilité. Ces dernières sont compétentes pour connaître des litiges liés à la remise d'un logement décent, à l'état des lieux, aux charges locatives et aux réparations, ou encore au niveau des loyers. Or, sur ces points, le bail mobilité est soumis au droit commun. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à étendre le recours aux commissions départementales de conciliation au bail mobilité.

la commission départementale de conciliation joue un rôle fondamental de médiateur et permet de rééquilibrer les rapports locataires-propriétaires. Elle peut être saisie par le propriétaire ou le locataire, et constitue ainsi un recours simple pour les locataires qui font face à des abus de la part de leurs propriétaires. Les CDC semblent ainsi essentielles dans le contexte du bail mobilité, bail qui par définition allège les contraintes légales prévues par la loi de 1989 qui s'imposent dans le cadre des baux traditionnels dans la mesure où celles-ci offrent un contrepoids à la perte de sécurité qu'engendre ce type de bail.

ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. La création du bail mobilité répond à la demande de location inférieure à un an, nécessaire pour les personnes amenées à changer fréquemment de résidence pour des raisons liées à leurs études ou à des motifs professionnels. Certes, ce nouveau bail présente des avantages pour le locataire, puisque le propriétaire ne pourra pas lui donner congé pendant cette période. Le dépôt de garantie n'est pas exigé, ce qui évitera bien des contentieux. Toutefois, que se passe-t-il si le locataire poursuit ses études supérieures, par exemple ? Tel que l'article est rédigé, il ne pourra rester dans le logement qu'à la seule condition que le propriétaire veuille bien conclure un bail meublé. Le présent amendement vise à permettre, au terme du contrat, la reconduction la reconduction du bail mobilité dans le respect des dispositifs applicables au bail meublé, afin que soit prise en compte la situation des locataires qui continuent de respecter les critères d'éligibilité. Il a également pour objectif d'éviter un recours excessif à ce type de bail, au détriment des autres locataires qui sont à la recherche d'une résidence.

remplissant les conditions requises pour la location du bail meublé pourrait, contre la volonté du bailleur, bénéficier automatiquement d'un nouveau bail meublé de droit commun. Il paraît donc préférable que, dans tous les cas, l'éventuel maintien dans les lieux

cela a été dit, être détourné de cet usage et utilisé pour contourner des baux plus sécurisants pour les locataires. Cela inquiète de nombreuses associations de défense des locataires et du droit au logement.

il y en a ! -, voire de marchands de sommeil. Nous proposons donc que l'interdiction concerne également le propriétaire. Autrement dit, un preneur à la fin du bail ne doit pas pouvoir signer un nouveau contrat de location mobilité pour le même logement ou avec le même propriétaire pour un autre bien lui appartenant. Il ne faut pas qu'un propriétaire puisse abusivement faire signer à un locataire une succession de baux temporaires, et fragiliser ainsi ses droits. l'avis de la commission ? Nous entendons vos inquiétudes quant à un possible détournement du dispositif par les marchands de sommeil, mais, juridiquement, on ne peut interdire la conclusion d'un bail entre un propriétaire et un locataire.

L'Assemblée nationale a exonéré le bail mobilité de cette obligation. La définition même du bail mobilité en fait un bail de courte durée ; il n'a donc pas vocation à servir pour une résidence principale, selon le Conseil d'État

l'avis de la commission ? Il convient, au contraire, de maintenir pour les logements objets d'un bail mobilité cette exonération de la procédure d'autorisation de changement d'usage. C'est un prérequis indispensable à la mise en oeuvre de ce nouveau bail. Supprimer cette disposition reviendrait à priver de tout à priver de tout effet utile l'adoption du bail mobilité. Le bail mobilité vise à répondre à des besoins de logement ; il ne soustrait donc aucun logement au marché du bail d'habitation. Son régime très encadré ne le rend pas plus attractif pour des investisseurs immobiliers

Cet amendement, qui a déjà été présenté à l'Assemblée nationale, vise à inscrire dans le code de la construction et de l'habitation un nouveau type de logement, en l'occurrence les résidences juniors. En

depuis la loi Égalité et citoyenneté, aucun décret n'a été pris, ce qui aboutit à une situation étrange dans laquelle il existe bien un statut pour les résidences universitaires, mais dont aucune résidence ne peut se prévaloir. Juridiquement, il n'y a donc aucune résidence universitaire aujourd'hui, alors qu'on estime le nombre de logements concernés entre 200 000 et 250 000.

favoriser l'accès au logement des ménages prioritaires, favoriser la mixité sociale, favoriser le parcours résidentiel des locataires de logements sociaux, et favoriser l'accueil des publics spécifiques.

Pour encadrer ces motivations, l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation précise que l'absence de lien avec la commune ne peut constituer, à lui seul, un motif de non-attribution d'un logement adapté aux besoins et capacités du demandeur. La préférence communale est un frein reconnu au logement des ménages en difficulté et un obstacle majeur à une plus grande mixité sociale. Cet amendement tend donc à totalement l'absence de lien avec la commune d'implantation du logement comme motif de non-attribution d'un logement social à un demandeur qui en a besoin. Quel est l'avis de la commission

Cette problématique a été largement explicitée dans l'excellent et récent rapport de nos collègues Michel Boutant et François Grosdidier, qui porte sur le malaise des forces de sécurité intérieure. Il nous faut envisager des solutions adaptées qui permettent à ces fonctionnaires d'accéder au logement. Concernant les logements sociaux des policiers, la situation est un peu particulière, puisque la préfecture de Paris a créé un bureau de logement, dont la mission est d'attribuer des logements conventionnés appartenant à des bailleurs privés. Or ce dispositif est aujourd'hui largement lacunaire. Mes chers collègues, ce dispositif est sous-utilisé puisque, sur les 3 200 policiers arrivés, seuls 400 y ont fait appel. Selon

très solennellement, monsieur le secrétaire d'État, pour que nos forces de l'ordre, qui assument des missions particulières et fondamentales pour notre République, trouvent les moyens d'accéder à un logement dans des conditions acceptables.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 35 du projet de loi. En effet, le dispositif de cet article prévoit d'élargir les missions de la commission d'attribution des logements, ou CAL, des bailleurs HLM. Ainsi, il est envisagé un réexamen tous les six ans de la situation des occupants d'un logement locatif social conventionné, en fonction de l'évolution de leur

Contrairement au Gouvernement, nous pensons que la démarche de changement de logement par le locataire doit être volontaire et non contrainte.

que cette disposition ne va pas dans le bon sens, elle peut être perçue comme une intrusion dans la situation familiale des occupants. En définitive, cet article porte une nouvelle fois atteinte au droit au maintien dans les lieux dans le parc social, d'où notre proposition de le supprimer

mais d'agir pour l'universalité du droit au logement et, donc, de l'accès au logement social. L'Union sociale de l'habitat dit souvent que le logement social est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est même le patrimoine commun de tous. Il convient donc de mobiliser tous les moyens pour agrandir ce parc public, en rassemblant des financements pour la construction, en utilisant les outils contre la vacance, ce qui facilitera l'utilisation d'outils permettant la transformation du parc privé en parc public public et favorisera la mixité sociale au sein même du parc HLM, conformément à notre vision universaliste du logement social. Si le logement social est le patrimoine de tous, alors tous doivent pouvoir y prétendre ! Ce relèvement du plafond aurait deux conséquences positives : la première, la plus fondamentale, serait de permettre à des personnes

La deuxième, qui se vérifie dans la pratique, serait de permettre aux maires bâtisseurs de répondre à un panel plus large de demandeurs et, donc, de faciliter les opérations de construction. Il arrive que des logements neufs restent vides, faute de locataires aux ressources suffisantes pour assumer un loyer. Ces logements relèvent certes du logement social, sont déjà largement inaccessibles pour le plus grand nombre. Le relèvement du plafond répond à notre vision généraliste du droit au logement et, donc, à notre volonté de renforcer la mixité sociale et urbaine.

Que dire de ces logements vides, faute de locataires répondant aux critères de ressources, qui sont extrêmement bas, puisqu'un couple de fonctionnaires débutants ne peut pas prétendre au logement social

important de logements sociaux restent vacants durant de longues périodes. Cela est notamment dû à la décroissance de l'activité dans ces zones et à l'abandon des commerces de proximité. Je ne vous ferai pas ici le laïus sur les services publics, mais ceux-ci ont eux aussi tendance à disparaître de nos zones rurales. Pourtant, nous restons convaincus qu'une approche favorisant l'accès au logement social et prenant en considération les disparités territoriales permettrait d'éviter le recours à de nouvelles exemptions aux objectifs de production fixés par la loi SRU,

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'avez constaté, nous avons dépassé minuit ... Je vous propose d'ouvrir la nuit et de prolonger nos travaux afin d'aller plus loin dans l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observations ? ... Il en est ainsi décidé.

de M. Raison a pour objet de permettre aux personnes dont l'habitat permanent est constitué d'une résidence mobile d'accéder plus facilement à des logements locatifs sociaux qui leur sont spécifiquement adaptés, en leur permettant de bénéficier du droit de réservation du préfet du préfet de département, à travers le contingent préfectoral défini aux articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation. Il y va de l'intérêt des personnes « sédentarisées » ou en voie de « sédentarisation », mais aussi de l'intérêt des collectivités locales qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas des outils pertinents en termes d'habitat pour répondre à cette évolution sociétale.

J'ai peut-être été trop rapide en me contentant de donner un avis favorable. Cet amendement prévoit que les logements du contingent préfectoral adaptés aux gens du voyage en voie de sédentarisation puissent bénéficier en priorité à ces personnes, les logements du contingent préfectoral adaptés aux gens du voyage en voie de sédentarisation puissent bénéficier en priorité à ces personnes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.

Pour que le système d'attribution soit plus juste et plus transparent, le contrôle des plafonds de ressources n'offre pas une donnée suffisamment précise et fine. En prenant systématiquement en compte le patrimoine, la commission pourra s'assurer que le locataire occupe bien son logement à titre de résidence principale. Cette disposition mettra un terme à des abus qui sont très largement minoritaires, mais qui suscitent de l'incompréhension et de la défiance dans la société française. Depuis 2016, l'État module déjà le montant des APL en fonction du patrimoine des allocataires. Rien ne justifie qu'il en soit autrement dans les commissions d'attribution. Quel est l'avis de la commission

le secrétaire d'État, mais, au sein de la CAL, le bailleur social est représenté. Je serais curieux de savoir combien de personnes sont expulsées

Pourtant, le rapport de la Cour des comptes publié en février 2017 dresse le constat d'un logement social qui manque en partie sa cible. En effet, environ la moitié des occupants ne serait ni défavorisée ni modeste, alors que la moitié des ménages situés sous le seuil de pauvreté est logée dans le parc privé. Continuer à produire davantage de logements sociaux constitue évidemment une partie de la réponse, mais cela prend du temps et les ménages en situation de précarité ne peuvent pas attendre. Le taux de mobilité dans le secteur social, qui n'est que de 9,7 %, doit évoluer. D'après le rapport, une augmentation d'un point de ce taux équivaudrait à la construction de 47 000 logements par an. pourquoi, pour améliorer la fluidité des parcours résidentiels, ainsi que pour s'assurer que les logements sont adaptés à la situation des ménages, le présent amendement vise à porter de six ans à trois ans la fréquence de l'examen périodique des conditions d'occupation des logements sociaux en zone tendue. Il rétablit en fait la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale. La durée de six ans ne reflète pas la réalité des changements de situation personnelle ou familiale, qui évolue rapidement, y compris en trois ans. Quel est l'avis de la commission

ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. La notion de sous-occupation constitue l'un des outils favorisant la mobilité du parc social. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 avait apporté un début de réponse, en modifiant les conditions d'application du surloyer de solidarité et du droit au maintien dans le logement, ainsi que la définition de la sous-occupation. La commission des affaires économiques du Sénat a souhaité revenir sur cette définition, en octroyant une pièce de plus : ainsi, le logement serait insuffisamment occupé, lorsqu'il comporte un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y résident, au lieu d'une pièce selon le droit en vigueur. Le présent amendement vise à supprimer cette modification de la définition de la sous-occupation afin de préserver la stabilité du droit en la matière et de ne pas entraver la mobilité au sein du parc social.

plus particulièrement les territoires situés en zone détendue, qui se trouvent dans l'obligation d'appliquer ces règles, alors que ni leur territoire ni l'occupation de leur parc ne le justifient. Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement

pour les locataires qui sont dans une situation de sous-occupation, de sur-occupation ou de revenus améliorés, en leur permettant de rester dans leur commune, sans être obligés de trouver

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement s'attaque à plusieurs problèmes liés au relogement. La loi de 1948 prévoit, pour les rares cas de relogement, des conditions qui ne sont pas assez sécurisantes pour le locataire. Dans le but d'instaurer une nécessaire équivalence pour le locataire, nous précisons donc que le nouveau logement doit correspondre à ses besoins familiaux et professionnels en termes de surface et de nombre de pièces. Nous précisons également que, sauf accord contraire du locataire, les dépendances- parking, cave ... -doivent être les mêmes à des tarifs identiques. Par ailleurs, pour faciliter l'exercice pénible et coûteux que représente un déménagement, nous proposons de créer une aide à la mobilité pour les locataires sous le régime de la loi de Nous précisons enfin que le dépôt de garantie ne peut excéder celui du logement précédent. Il semble nécessaire que ces conditions soient remplies pour que l'esprit de la loi en matière de relogement soit respecté. Rappelons qu'un relogement peut remettre en cause l'équilibre entier d'une vie ! La loi doit éviter qu'il ne devienne un calvaire. Quel est l'avis de la commission

malheureusement, plus petits que ceux d'avant et que ces cas de relogement sont souvent l'occasion d'octroyer un logement plus adapté à la personne. Les conditions d'une aide à la mobilité, prise en charge par l'organisme chargé de l'opération d'urbanisme, sont déjà prévues dans le code de la construction et de l'habitation,

Cela implique d'orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d'urgence. Or, ces dispositifs sont plus que jamais saturés. Le parc des hébergements d'urgence peine à jouer son rôle de tremplin vers le logement.

seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'autre conjoint a fait la demande d'un titre de séjour ou d'une demande d'asile et se trouve dans l'attente d'une décision définitive relative à son droit au séjour. C'est pourquoi nous proposons dans cet amendement de distinguer le titulaire du bail, dont le séjour est régulier, du conjoint- époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer. Cette possibilité permettrait à des ménages d'accélérer leur sortie des dispositifs d'hébergement d'urgence, d'autant que la loi

est inconditionnel, ce n'est pas le cas du logement social. L'avis est donc défavorable

Pourquoi ? À notre sens, la généralisation de ce dispositif pourrait en pratique se révéler très contraignante en empêchant de s'adapter aux réalités locales et de répondre aux situations d'urgence. Je souligne également que, lors de la conférence de consensus sur le logement, un certain nombre de participants s'étaient élevés contre cette généralisation du système de cotation. La commission des affaires économiques a souhaité en rester au droit actuel, c'est-à-dire que le système demeure, mais qu'il soit facultatif. Il laisse donc bien la possibilité aux EPCI de décider

L'article 37 tend à simplifier le dispositif d'attribution de logements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Outre le fait que ces quartiers sont souvent partie intégrante de communes dont la population et le maillage urbain n'ont qu'assez peu à voir avec les villes résidentielles et touristiques de certaines agglomérations favorisées, il importe d'éviter qu'ils ne soient, plus encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, victimes des processus ségrégatifs développés depuis un peu plus de quarante La première attaque, qu'on le veuille ou non, fut portée par le gouvernement Barre qui, en suspendant le mode de financement ordinaire des HLM pour développer le financement PLA, ... Ouh là ! Ça fait du bien à cette heure-ci de revenir un peu en arrière le financement PLA et en créant les aides personnelles au logement, a été à l'origine d'une croissance constante de la dépense publique pour compenser les effets pervers du marché. La loi Méhaignerie, qui prétendait lutter contre l'inertie de la loi de décembre 1948, a conduit à la marchandisation du logement, la constitution et la croissance des copropriétés dégradées, la flambée des loyers du secteur privé et la segmentation du marché, comme des aspirants locataires. Le « pognon de dingue » que la France dépense pour couvrir les désordres du marché, monsieur le secrétaire d'État, il vient de là, et votre texte, malheureusement, risque fort d'y contribuer plus encore. il convient d'éviter aux quartiers prioritaires de la politique de la ville de devenir, plus encore qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui, des « ghettos de la misère », aussi lépreux que peuvent être rutilants les « ghettos du gotha », édifiés parfois à quelques kilomètres des premiers. Si l'article 37 entend laisser libre cours à l'appréciation des acteurs locaux en matière de logement, laissons-leur donc la possibilité d'attribuer un certain nombre de logements à des personnes dont les ressources pourraient dépasser les plafonds retenus.

La commission souhaite avoir l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques. Sur la première proposition, la rédaction issue de l'Assemblée nationale me semblait un bon compromis, car cette pré-CAL ne pourra être réunie que sur demande du maire de la commune où se trouve un QPV. Sur la seconde proposition, actuellement, les dispositions légales et réglementaires permettent déjà au préfet de fixer des plafonds de ressources dérogatoires, par immeuble ou par secteur dans les QPV, pour favoriser la mixité sociale. Il en est de même pour un immeuble ou un ensemble immobilier occupé à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des APL. Je m'interroge : ne risque-t-on pas de créer des

que « le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources » -donc aux plafonds de ressources -, s'il s'agit de « faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, pour permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers » mentionnés dans un autre article. Cela répond précisément au souhait

Cet amendement concerne les conditions dans lesquelles l'Association foncière logement, l'AFL, peut céder ses logements, ce qu'elle a l'obligation de faire, je vous le rappelle, puisqu'elle se constitue un patrimoine

entre les principales organisations représentatives de bailleurs et celles des locataires pour traiter des difficultés suscitées par la délivrance de congés pour vente aux locataires. L'article 1.1 de l'accord

occupation. Or l'AFL ne délivre pas de congés pour vente et maintient ses locataires en place dans les mêmes conditions de location que dans le cas où ils ne souhaitent pas se porter acquéreurs. Pour autant, même en l'absence de délivrance d'un congé pour vendre, il ressort que les obligations d'information du locataire qui a reçu une offre d'achat de son logement sont les mêmes que celles bénéficiant au locataire qui réceptionne un congé pour vendre. La mise en place des accords collectifs des locataires se révèle extrêmement contraignante pour l'AFL et contre-productive pour la mise en oeuvre du plan de cession, notamment au regard des contraintes administratives et des délais à respecter. Par ailleurs, la mise en application des accords collectifs se justifie d'autant moins que l'AFL s'engage à apporter une information totale et complète aux locataires, futurs accédants, sur la résidence, le logement, l'environnement,

Si j'ai bien compris, votre amendement vise à exclure une entité qui s'appelle l'AFL, l'Association foncière logement, des accords collectifs de 2005.

à la découpe, par lots de cinq logements. Actuellement, l'article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la cession de logements conventionnés à l'APL du groupe Action Logement ne donne pas lieu à un congé pour vente.

les caractéristiques de l'AFL par rapport aux autres entités soumises à l'accord collectif de 2005 ne me semblent pas justifier d'écarter l'AFL de cet accord collectif de 2005. Si je n'ai pas été suffisamment convaincant et précis, je veux bien en rediscuter un matin de bonne heure avec vous. Je pense que l'on était à peu près sur la même longueur d'onde, mais le problème posé à Action Logement vient du fait que l'AFL ne vend pas en ayant libéré le logement,

de remettre en cause, à terme, les modalités de financement, dans la mesure où le réservataire ne connaîtra pas à l'avance la localisation et la qualité des logements qui lui seront proposés. Ensuite, la commission a maintenu la possibilité de déroger au taux de 25 % d'attributions de logements sociaux à des personnes appartenant au quartile des personnes ayant les revenus les plus faibles, dans le cadre des orientations en matière d'attribution adoptées par la conférence intercommunale du logement. Elle a également précisé que, pour l'application de l'obligation d'attribuer 25 % de logements sociaux à des personnes appartenant au quartile des personnes aux revenus les plus modestes, en dehors des quartiers les zones urbaines sensibles seront assimilées à ces quartiers pendant une durée de six ans. Il s'agit ainsi de ne pas fragiliser des quartiers qui viennent juste de sortir de la géographie prioritaire en y envoyant de nouveau des personnes figurant parmi les plus pauvres. Pour l'application de cette même obligation, elle a enfin relevé le seuil du premier au deuxième quartile pour ne pas pénaliser les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Certes, ces modifications sont profondes, comme vous l'avez souligné, mais je pense qu'elles vont vraiment dans le sens de la diversité des territoires. Surtout, elles ont pour but de laisser la main aux maires, pour qu'ils puissent véritablement décider des personnes qu'il y a lieu de loger, y compris dans des territoires tout

du Gouvernement, pour revenir au premier quartile et intégrer les handicapés, ce qui nous permettra, je pense, de rééquilibrer globalement le travail fait par la commission. Même si

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a instauré des obligations de mixité sociale pour l'attribution de logements sociaux. Ainsi, 25 % des attributions annuelles en dehors des quartiers prioritaires de la ville doivent bénéficier au premier quartile des ménages les plus modestes. La conférence intercommunale du logement peut toutefois adapter ce taux en fonction de la situation locale. Cette possibilité nuit à l'efficacité de la mesure. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui rend obligatoire l'application du taux de 25 %. La portée de cette obligation a également été amoindrie avec l'introduction, en commission, du deuxième quartile des ménages les plus modestes dans le dispositif. Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi adoptées par l'Assemblée nationale

dans certains quartiers de la politique de la ville, a été supprimée en commission des affaires économiques. Avec cet amendement, nous proposons de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale, qui prévoit qu'au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient à des demandeurs dont les revenus sont supérieurs au seuil du premier quartile.

Ainsi, la ville de Nanterre, dont le taux de logements sociaux atteint les 56 %, a relogé, en 2017, 248 ménages prioritaires, dont 198 personnes éligibles au DALO et 50 familles au titre des publics prioritaire, dépassant ainsi largement les objectifs fixés par la préfecture. Cette proportion ne cesse de croître et pénalise au final les communes qui ont fourni d'importants efforts dans ce domaine. Il est à noter, en outre, que le relogement de ces publics intervient dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui va à l'encontre de la stratégie souhaitée par le Gouvernement, qu'a présentée le 22 mai dernier le Président de la République. Il apparaît donc nécessaire de prévoir des niveaux d'attribution différenciés pour les communes dont le taux de logements sociaux est compris entre 40 % et 50 % ou dépasse les 50 %.

Des poursuites et des recours indemnitaires sont engagés parce que l'État ne reloge pas dans les délais raisonnables les bénéficiaires du DALO. Par ailleurs, une évaluation a montré que la délégation n'a pas fonctionné comme elle aurait dû. C'est pourquoi la loi Égalité et citoyenneté a supprimé la délégation des droits de réservation du préfet. commission des affaires économiques a quant à elle rétabli la possibilité, pour le préfet, de déléguer son contingent. Dans la même logique que nos amendements précédents, nous proposons donc de limiter cette délégation aux seules communes disposant sur leur territoire de plus de 35 % de logements sociaux et d'un quartier prioritaire de la ville.

pour désigner de nouveaux candidats. Dans ces quartiers, en cas de difficulté de remise en location, le maire est en effet le mieux à même d'appréhender les différents enjeux d'équilibre d'occupation sociale du territoire.

Le bailleur peut, le cas échéant, vouloir vérifier des informations transmises par le candidat locataire en cas de pièces incohérentes ou douteuses. Les agents de gestion pourraient conclure trop vite à une fraude ou à la production de faux, ce qui inclut une qualification pénale et donc un risque, pour le bailleur, de se voir reprocher le délit de dénonciation calomnieuse. À l'inverse, en cas de fraude avérée, le bailleur pourrait se voir reprocher de ne pas avoir suffisamment vérifié les pièces du dossier. Pourrait-il tout de même agir en justice et demander la nullité du bail pour dol ? pourrait-elle lui reprocher son inaction ? Il serait véritablement plus simple pour les bailleurs de pouvoir exiger du candidat lui-même la justification ou l'explication des cas d'incohérence ou d'irrégularité